vote. Monsieur le président, lors du scrutin n° 44 sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2020, M. Alain Bertrand a été enregistré comme s'abstenant, alors qu'il souhaitait voter pour.

Mes chers collègues, je veux saluer en votre nom la présence, dans notre tribune d'honneur, d'une délégation de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, conduite par M. Andrés Castro Alegria, vice-président du groupe d'amitié Cuba-France, président de la commission de l'éducation, de la culture, de la science, de la technologie et de l'environnement. La délégation est accompagnée par notre collègue Hélène Conway-Mouret, vice-présidente du Sénat et présidente du groupe d'amitié France-Caraïbes. Nous entretenons des relations très constructives avec nos homologues de l'Assemblée nationale cubaine. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique du renforcement des relations entre nos deux pays, en particulier sur le plan politique, mais également dans le domaine scientifique et universitaire, ainsi qu'en témoigne le développement d'accords récents de coopération universitaire. En votre nom à tous, permettez-moi, mes chers collègues, de souhaiter à nos homologues de l'Assemblée nationale de Cuba la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour. L'ordre du jour appelle la suite

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » (et article 73

dans le cadre de l'examen de cette mission, je voudrais d'abord exprimer notre respect et notre reconnaissance aux treize militaires décédés lundi soir, au Mali, en adressant nos sincères condoléances à leurs familles durement éprouvées, ainsi qu'à notre collègue Jean-Marie Bockel. Je voudrais associer à cet hommage nos militaires, nos gendarmes, nos policiers, nos sapeurs-pompiers, l'ensemble des forces de sécurité qui risquent leur vie au quotidien pour la sécurité des personnes et des biens et qui luttent aussi contre le terrorisme.

Ces réductions de crédits résultent de faits démographiques malheureusement implacables, mais aussi d'un choix budgétaire qui jure avec les témoignages de considération adressés au monde combattant qui mérite respect et reconnaissance. Le rapport « constant » qui conditionne l'indexation des valeurs des pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant conduit au gel de ces allocations et donc à leur baisse en

et des élus. Le Président de la République a pris des engagements pour assurer un État de proximité. La restructuration de l'ONAC-VG obligera-t-elle les anciens combattants et les pupilles de la Nation à à s'adresser aux maisons France services pour accéder aux accompagnements qui leur sont si nécessaires ? Les missions de l'ONAC-VG ont fait l'objet d'une diversification constante. La structure rencontre des difficultés significatives pour les mener à bien, notamment le traitement des demandes, les programmes de rénovation des lieux de mémoire et l'action sociale, laquelle reste aussi l'une des priorités de l'Office. Parmi nos inquiétudes figure la répétition répétition de certains constats relatifs à la JDC. Trop de jeunes encore manquent à la fréquentation de ce rendez-vous avec nos armées. Un motif de satisfaction est à relever dans la revalorisation

d'information. On ne retrouve pas, dans le projet de budget, les moyens d'une « CIVS augmentée », plus proactive et mieux capable d'achever un processus de réparation. réparation. J'appelle solennellement votre attention, madame la secrétaire d'État, et celle du Premier ministre, sur l'impérieuse nécessité de traiter convenablement le dossier des parts réservées qui laissent une dette de réparation de plusieurs dizaines de millions d'euros encore impayée. La commission des finances, attentive aux sollicitations légitimes du monde combattant, et lui ayant clairement apporté tout son soutien, recommande l'adoption des crédits de la mission. La parole est à M.

Nous partageons profondément leur douleur et leur disons toute notre reconnaissance pour l'engagement sans faille des leurs au service de la France pour assurer notre sécurité. C'est donc avec une grande tristesse que nous examinons ce matin les crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ». Ces crédits baisseront en 2020, comme c'est le cas chaque année. Cette baisse ne peut être imputée à des mesures d'économies ou à une dégradation du traitement des anciens combattants, puisqu'elle résulte largement de la disparition progressive de ceux qui ont qui ont servi au cours des grands conflits du XX siècle, alors que les « jeunes » générations d'anciens combattants, si je peux m'exprimer ainsi, sont nettement moins nombreuses. Les économies découlant de cette évolution démographique permettent parfois d'améliorer les dispositifs existants. L'an dernier, la carte du combattant a été accordée aux soldats ayant servi en Algérie entre 1962 et 1964. Cette année, un geste est fait en faveur des veuves de grands invalides. Ces mesures sont toutefois très marginales. Pourtant, certaines revendications du monde combattant mériteraient d'être étudiées avec bienveillance par le Gouvernement. Je pense notamment à la revalorisation du point d'indice des pensions militaires d'invalidité qui a évolué moins vite que l'inflation au cours des dernières années. La réunion d'une commission tripartite nous est promise pour 2020. Nous l'attendons avec impatience, madame la secrétaire d'État. Sans préjuger des recommandations qu'elle pourrait formuler, il me semble qu'une règle simple d'indexation sur l'inflation pourrait être posée. D'autres demandes existent, plus ou moins légitimes et plus ou moins prioritaires ; certaines font l'objet d'amendements que nous étudierons tout à l'heure. Si la baisse des dépenses liées à la reconnaissance et à la réparation est compréhensible, il aurait été souhaitable que la disparition des derniers témoins des grands conflits s'accompagne d'un effort financier accru en faveur du soutien aux projets éducatifs et mémoriels. Nous savons tous combien la transmission de la mémoire, surtout s'agissant des heures difficiles de notre histoire nationale, est nécessaire à la formation des citoyens de demain. Par ailleurs, les élus de terrains que nous sommes tous sont attentifs au maintien du maillage territorial assuré par les offices départementaux de l'ONAC-VG. Je crois savoir que vous y êtes également attachée, madame la secrétaire mais que des positions différentes peuvent exister. Je souhaiterais enfin dire un mot du prélèvement opéré sur la trésorerie de l'ONAC-VG. Cette mesure peut paraître acceptable en 2020. En effet, l'excédent de cet opérateur apparaît excessif au regard des objectifs de bonne gestion budgétaire. Toutefois, madame la secrétaire d'État, nous espérons que vous saurez obtenir, l'année prochaine, les arbitrages nécessaires pour que vous soient accordés les crédits dont vous vous passez cette année. La commission des affaires sociales a donc donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission pour 2020 et sera vigilante, l'année prochaine, au rétablissement des crédits consacrés aux dépenses mises cette année à la charge de l'ONAC-VG.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, j'avais envisagé d'entamer mon propos en évoquant le cent unième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, cette guerre terrible qui a marqué les mémoires et changé le monde. J'avais envisagé de rendre hommage à l'ensemble de nos vétérans de métropole et d'outre-mer et de saluer la mémoire de celles et ceux qui ont disparu et l'actualité nous a ramenés à une autre réalité. Nous inscrirons bientôt sur le monument aux morts en opérations extérieures (OPEX), inauguré récemment par le Président de la République, treize nouveaux noms : treize noms de soldats de la force Barkhane engagés au Sahel pour lutter contre le terrorisme ; treize incarnations de ces soldats

La reconnaissance de la Nation ne doit pas seulement se traduire dans des mots. Elle doit s'incarner dans des actions au bénéfice de nos soldats et de leurs familles. Dans le souci de réaffirmation des valeurs et de reconnaissance des combattants, j'avais déposé une proposition de loi pour que les militaires ayant combattu pour la France aient droit à une draperie tricolore sur leur cercueil. Les militaires doivent accomplir des démarches administratives lourdes, et parfois complexes, pour obtenir la carte du combattant et les avantages qu'elle octroie- dont la draperie tricolore. Il nous semble pourtant que les militaires ne doivent pas avoir à quémander ce qui leur revient de droit. C'est la Nation qui doit s'assurer qu'ils obtiennent ce à quoi ils ont droit. Cette proposition de loi n'a malheureusement pas fait l'unanimité. Le groupe Les Indépendants a néanmoins continué à travailler pour faire évoluer le droit en ce sens. Et nous sommes parvenus à obtenir un engagement écrit de Mme Mme la secrétaire d'État, que je remercie. Les militaires, dès leur retour d'OPEX, seront désormais épaulés par leur unité pour remplir ces demandes et chaque militaire éligible à cette carte du combattant en sera individuellement informé. Voilà des avancées concrètes pour nos soldats. Il en faut d'autres. Le budget que nous examinons aujourd'hui doit contribuer à l'amélioration de la vie des anciens combattants malgré la diminution des crédits confirmée pour 2020. Cette évolution s'explique notamment par la diminution structurelle du nombre de bénéficiaires des différents dispositifs. Nous veillerons naturellement à ce que cette diminution tendancielle ne représente pas un déclin de la reconnaissance de la Nation ni des conditions de vie des bénéficiaires. Nous tenons à saluer l'amélioration annoncée de la réversion de la pension militaire d'invalidité versée aux conjoints survivants de grands invalides de guerre. Des pistes d'amélioration demeurent. Nous regrettons que ce budget ne soit pas plus ambitieux, notamment en ce qui concerne la revalorisation des pensions militaires d'invalidité. Nous espérons que les résultats de la concertation, qui reste en suspens, aboutiront à l'amélioration de la situation des bénéficiaires. Le budget poursuit également une action à destination de la jeunesse. Les objectifs en sont louables et nous les partageons pleinement. Il s'agit notamment de transmettre aux jeunes les valeurs de la République. Mais la réalisation nous interroge : les programmes se multiplient et leur coût s'alourdit. Le service national universel (SNU) engagera probablement autour de 50 millions d'euros- si ce n'est plus -, bien au-delà du chiffrage prévisionnel. En outre, est-ce à l'armée, qui a déjà fort à faire par ailleurs, d'assurer la formation citoyenne de nos jeunes Français ? Elle en sera probablement chargée, faute d'une alternative crédible susceptible d'accomplir cette mission. Le budget que nous examinons est lourd de sens. Il touche à l'un des piliers de la Nation, aux valeurs qui sont le socle de l'engagement, de l'acceptation du risque et du sacrifice dont font preuve nos soldats. Il nous faut garder en tête ces enjeux et nous montrer à la hauteur. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, servir la France sans relâche, malgré les difficultés, malgré l'ennemi, c'était la raison d'être de nos treize militaires décédés voilà deux jours au Mali. Je veux tout d'abord leur rendre hommage et adresser à leurs familles mon total soutien et mes pensées les plus émues. La guerre, n'est pas l'acceptation du risque. Ce n'est pas l'acceptation du combat. C'est à certaines heures, pour le combattant, l'acceptation pure simple de la mort ». Ces mots de Saint-Exupéry nous rappellent ce que représente, pour nos combattants d'hier et d'aujourd'hui, le fait de servir notre nation au nom de valeurs qui transcendent leurs propres intérêts, leurs propres sentiments, voire leur destin personnel. Pour certains d'entre eux cet engagement a parfois pris la forme, ultime, du sacrifice. À ces femmes et à ces hommes, à ces mères et à ces pères, à ces héros, la République tout entière est reconnaissante. Aussi, cette action de mémoire, nous la leur devons. Plus qu'un devoir, elle est une nécessité. Un peuple qui se détournerait de son passé serait un peuple sans âme, en perte de direction. En déterminant la reconnaissance de l'État et en fixant la politique de mémoire, cette mission budgétaire demeure importante. Elle est au croisement de l'histoire passée, présente et future. En sommes, le budget alloué dans le cadre de ce projet de loi de finances s'inscrit dans une trajectoire baissière.

Quant au service militaire volontaire (SMV), je ne peux qu'insister sur son importance : plusieurs fois par an, sur la base aérienne de Brétigny-sur-Orge, je rencontre des jeunes particulièrement motivés. Ils ont tous connu des parcours difficiles, mais une seconde chance leur est offerte par la société. Le taux de réussite demeure très satisfaisant.

C'est là une très belle initiative qui rend hommage aux combattants ayant payé un lourd tribut au nom de la liberté. Cette cérémonie était solennelle et empreinte d'une émotion particulière pour les conjoints et les enfants présents. Dans son intervention, le Président la République a rendu hommage aux soldats morts au combat. Il a aussi rappelé aux familles que la République ne les oubliait pas, qu'elle était à leurs côtés, malgré la peine et la souffrance. Dans ce prolongement, il serait souhaitable que le Gouvernement s'engage à honorer plus régulièrement la mémoire des dissidents d'outre-mer qui, par attachement aux valeurs républicaines, avaient décidé de rejoindre la métropole dans le seul but de sauver la patrie et de vaincre l'ennemi. Cette autre armée de l'ombre met décidément bien du temps à entrer dans la lumière ». N'oublions pas leur courage. À ce stade de mes propos, il m'est impossible de ne pas penser aux nombreux porte-drapeaux et bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui oeuvrent dans nos territoires pour la réussite des commémorations. Sans eux, nos cérémonies n'auraient pas le même sens. Madame la secrétaire d'État, nous devons penser collectivement à la manière dont notre pays peut leur témoigner sa reconnaissance. Le lien intergénérationnel, c'est le défi d'aujourd'hui.

Nous regrettons la baisse des crédits provisionnés pour les allocations de reconnaissance aux rapatriés qui me semble profondément injuste. Ils ont aussi été aux côtés de la France ; nous leur devons une juste reconnaissance. La majoration des pensions militaires d'invalidité perçues par les conjoints survivants de grands invalides constitue une bonne nouvelle, même si, eu égard au nombre de bénéficiaires potentiels, l'impact budgétaire demeure très limité. limité. Il faut mener une réflexion plus générale sur les mesures en faveur des aidants, aussi bien sur leur accompagnement que sur le répit. En outre, année après année, nous évoquons la nécessité de mieux reconnaître l'engagement des personnels de l'opération Sentinelle. Les réservistes, souvent rappelés pour des périodes courtes, devraient bénéficier du titre de reconnaissance de la Nation. Leur attribuer ce droit serait une mesure de justice et d'égalité. Pour terminer sur ce programme, nous notons aussi la baisse de 12,5 millions d'euros des dotations pour l'ONAC-VG. Nous restons très attachés à son rôle. Il est souhaitable que nous restions vigilants sur son avenir. À cet égard, ne conviendrait-il pas de renommer l'ONAC-VG en Office national des « combattants » et victimes de guerre plutôt que des « anciens combattants »

Enfin, les dotations du programme 158 baissent également de 12 %, principalement du fait de la chute des moyens consacrés à la réparation des spoliations antisémites. C'est considérable. Mes chers collègues, au-delà même de ce débat budgétaire, soyons toujours vigilants face à la haine humaine, quel que soit son visage ou son message. Si elle tend parfois à progresser sournoisement, elle n'a pas sa place dans notre République. L'histoire nous l'a déjà démontré. Les Français, de toute confession ou origine, forment un seul bloc, celui de la communauté nationale.

et votre sens de l'écoute. Je vous sais pleinement mobilisée sur ces sujets, comme vous l'avez été pour la carte du combattant attribuée aux soldats présents en Algérie entre 1962 et 1964. Aussi, le groupe Union Centriste votera les crédits de cette mission, en espérant des évolutions futures. La parole

soit une baisse de 6,2 %. Soulignons que la mission avait déjà perdu 150 millions d'euros en 2019 ... Le Gouvernement rappelle, comme chaque année, que cette diminution de crédits serait liée à la baisse structurelle des effectifs du monde combattant. Or les marges de manoeuvre libérées par la diminution naturelle du nombre d'anciens combattants et de leurs ayants droit sont estimées à 100 millions d'euros par an. Celles qui sont dégagées cette année ne donnent malheureusement pas lieu à des mesures de revalorisation. Ainsi, le programme 169 qui regroupe la majeure partie des crédits de la mission pour financer les témoignages de reconnaissance de la Nation envers ses anciens combattants, avec près de 2 milliards d'euros, enregistre une baisse de dotation de 5,8 %. pour financer les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et d'autres interventions sont donc réduites. Pour 2020, la seule mesure d'extension des droits concerne les conjoints survivants des anciens combattants grands invalides, avec un impact limité

Nous présenterons un amendement visant à demander un rapport au Gouvernement sur la revalorisation du point de pension militaire d'invalidité et sur les solutions destinées à compenser les retards l'ayant affectée. L'action en faveur des rapatriés représente 0,9 % des crédits du programme 169, soit 18,7 millions d'euros contre 23,2 millions en 2019. L'allocation de reconnaissance, instituée par loi de 2005, constitue la principale dépense avec 88 % des crédits. Nous avons souhaité présenter un amendement visant à résoudre la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. En effet, 25 personnes ne bénéficient toujours pas de l'allocation de reconnaissance. Il est temps de réparer une injustice.

La diminution des moyens de l'Office a malheureusement des répercussions au niveau local. Ainsi, 42 emplois sont supprimés en 2020, dont 25 dans les services départementaux. Il est pourtant impératif de conserver le maillage territorial de l'Office, au risque de réduire la présence de proximité et de dégrader la qualité des services fournis aux personnes. En outre, la dématérialisation ne doit pas être le prétexte à de nouvelles économies au détriment de l'accompagnement du monde combattant. Enfin, l'une des nouvelles missions de l'ONAC-VG est la prise en charge économique et financière des victimes du terrorisme. Cette mission va malheureusement- mais certainement -monter en charge dans les prochaines années, nouvel argument en faveur d'une augmentation du budget de l'Office. Évoquons maintenant le programme 158, qui finance différentes indemnités accordées aux victimes d'actes de barbarie et de persécution commis pendant l'Occupation. ce programme sont en baisse de 11,7 % ; cette baisse pose de sérieux problèmes. En effet, l'an dernier, le Sénat avait souhaité l'extension de l'indemnisation des orphelins de victimes d'actes de barbarie, mais le budget pour 2020 ne le permet malheureusement pas.

Pourquoi cette baisse ? Elle s'explique certes par l'achèvement du mémorial consacré aux soldats morts pour la France en opérations extérieures et par la fin de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale ; mais nous estimons que les actions de mémoire ne devraient pas être à ce point dépendantes de commémorations exceptionnelles. ce budget se doit de faire vivre la mémoire ! À ce stade de mon intervention, je veux évoquer un sujet qui me préoccupe tout particulièrement : celui de la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, plus grande nécropole militaire française

Ces chiffres rendent incompréhensible le retard pris dans le financement des infrastructures d'accueil du site. Par exemple, le manque de sanitaires dignes de ce nom dans ce haut lieu de mémoire est scandaleux ! Je souhaite donc, madame la secrétaire d'État, vous interroger de nouveau aujourd'hui : ces travaux tant attendus vont-ils enfin

Cette réalité d'hier fait tristement écho, aujourd'hui, au drame qui vient de se dérouler au Mali. En pleine opération de combat, treize hommes, militaires aguerris, sont allés au bout de leur engagement pour servir leur pays. au nom du groupe du RDSE, rendre hommage à leur courage et adresser toutes nos pensées aux familles touchées, avec une attention particulière pour notre collègue Jean-Marie Bockel. Mes chers collègues, je commencerai par évoquer les moyens consacrés à la reconnaissance et à la réparation en faveur du monde combattant, qui mobilisent l'essentiel des crédits alloués à cette mission. Comme chaque année, ils enregistrent une diminution. La baisse du nombre d'allocataires des pensions d'anciens combattants ne devrait-elle pas nous conduire à profiter de la marge budgétaire naturellement dégagée pour enrichir le droit à réparation ? Il nous faudrait notamment revaloriser le point d'indice de la pension militaire d'invalidité. Du fait de son quasi-gel, la PMI individuelle moyenne aura décru de près de 300 euros entre 2018 et 2020.

Cependant, comme l'a souligné M. le rapporteur spécial, ce dispositif ne profitera malheureusement qu'à 461 personnes ; peut-être faudrait-il, à l'avenir, élargir son bénéfice à d'autres aidants. aidants. Au sein de ce même programme, je tiens à dire l'inquiétude que suscite l'actuelle restructuration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La subvention qui lui est allouée pour charges de service public diminue de 12 millions d'euros, à mettre en rapport avec une baisse de 3,7 % de ses effectifs, autant dire une véritable ponction pour l'opérateur. Cette solution n'est ni durable ni souhaitable. Rappelons que l'Office est le principal acteur de cette mission et qu'il est perçu, grâce à son maillage territorial, comme la « maison des combattants ». Son action diffuse et essentielle au plus près du monde combattant légitime le maintien de sa trésorerie. En effet, si le nombre global des anciens combattants diminue, ses missions s'élargit, comme ses catégories de ressortissants, des militaires envoyés en opération extérieure aux victimes d'attentats terroristes. J'ajoute que cet office est le référent privilégié des 8 000 associations d'anciens combattants et qu'il devra demain préserver leur patrimoine mémoriel pour en pérenniser la transmission. Il assure l'entretien des hauts lieux de la mémoire nationale et des sépultures, avec l'aide du Souvenir français il accueille le public sur les lieux de mémoire, reçoit les enfants de harkis ou encore participe aux modules « mémoire » du service national universel. C'est pourquoi la restructuration en cours doit être envisagée non comme une réduction, mais plutôt comme une réinvention de l'Office. Je veux dire aussi quelques mots du programme « Liens entre la Nation et son armée », qui nous est cher La baisse des crédits qu'emporte la fin du cycle des commémorations est compréhensible, mais je regrette les conséquences qu'elle aura sur l'entretien des sépultures et autres lieux de mémoire, que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre devra compenser par un prélèvement sur sa trésorerie. Dans ce domaine aussi, l'effort doit être constant, car il incarne l'hommage indéfectible rendu par la France à ceux de ses enfants qui sont morts pour elle. Il en va de même pour les monuments aux morts, et nous ne pouvons que saluer l'inauguration du monument aux morts en OPEX érigé dans le jardin Eugénie-Djendi, le 11 novembre dernier. Enfin, s'agissant des crédits du programme relatif à l'indemnisation des victimes des spoliations et persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale, ils accusent une diminution de 12 %. Là aussi, si cette contraction est structurelle, assurons-nous, près de vingt ans après la création de ce dispositif de réparation, que l'indemnisation soit la plus large possible. Dans un souci d'équité, mon groupe souhaiterait ainsi étendre le dispositif de réparation aux pupilles de la Nation dont les parents résistants sont morts pour la France les armes à la main.

ses armées. La mission interministérielle « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » rassemble les crédits consacrés à l'adhésion de la population aux efforts en faveur de la défense et de la sécurité nationales, depuis la fin de la conscription en 1997. Avec un total de 2,16 milliards d'euros en crédits de paiement pour 2020, le budget de cette mission est en baisse, alors même que les dispositions existantes sont maintenues. Cette baisse ne traduit aucun désengagement politique. Elle est seulement la conséquence mécanique d'une décroissance démographique naturelle du nombre de bénéficiaires.

Dans ces conditions, la diminution de 142 millions d'euros de la dotation budgétaire, cette année, paraît naturelle quand on sait que 94 % des montants alloués à la mission correspondent à des aides économiques et financières versées aux anciens combattants et aux victimes de guerre. sommes appelés à nous prononcer est équilibré et ambitieux, pour trois raisons. Tout d'abord, il traduit la priorité donnée au maintien des revenus des 2,4 millions de bénéficiaires, avec 912 millions d'euros de pensions militaires d'invalidité et 660 millions d'euros de pensions de retraite en faveur des anciens combattants. Cette priorité s'accompagne de la consolidation des droits des pensionnés, selon une approche renouvelée de la reconnaissance que leur Les pensions militaires des conjoints de grands invalides qui ont renoncé à toute activité pendant plus de quinze ans pour prodiguer des soins constants à leur conjoint invalide sont revalorisées. En concertation avec les associations, le Gouvernement avait tenu à reconnaître l'engagement des oubliés de la guerre d'Algérie ; cette reconnaissance concerne potentiellement 50 000 militaires ayant combattu en Algérie entre juillet 1962 et juillet 1964.

dont 13 millions d'euros d'investissements pour la création d'un pôle de réhabilitation post-traumatique. Enfin, les auteurs de ce budget pensent à l'avenir volonté de rationaliser l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, afin d'améliorer son efficacité dans l'exercice de ses missions d'assistance tout en maintenant une présence locale assurée par les offices départementaux des anciens combattants. Madame la secrétaire d'État, ce budget est donc un budget des engagements tenus. Permettez-moi de vous en remercier. Pour cette raison, le groupe La République En Marche votera les crédits de cette mission marquée par l'équité, la reconnaissance et le profond respect envers ceux qui ont consacré leur vie à notre pays. La

Faire des économies en spéculant sur la baisse démographique naturelle du nombre de bénéficiaires des pensions et de la retraite du combattant n'honore pas le Gouvernement.

dit, alors que nous pourrions satisfaire les droits à réparation du monde combattant depuis des années, le Gouvernement fait fondre le budget de la mission « Anciens combattants » et laisse ainsi dans la précarité des femmes et des hommes qui ont permis à la France d'être la terre de paix qu'elle est. qui leur est dû, nous devons le préserver, à l'heure où la haine, les extrémismes, les intégrismes et le rejet de l'autre sont toujours plus exacerbés, en France et en Europe.

de traçabilité, je note que le décret de juillet 2010 prévoit que « [l]'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés Tout le problème réside dans cette dernière phrase, puisque l'on dénombre aujourd'hui 135 unités combattantes pour lesquelles la France ne dispose plus de l'historique des opérations.

lieu, comment traiter de réparation sans évoquer le rapport constant ? Avec la réforme du rapport constant, en 2005, la valeur du point de PMI a été révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice Insee des traitements bruts de la fonction publique d'État.

du projet de loi de finances pour 2020 coïncide avec l'augmentation de 0,83 % de la valeur du point de PMI, le retard demeure de 7,13 %.

Morts d'hier, morts d'aujourd'hui, la France doit être digne de leur mémoire. Le cimetière et la basilique de Notre-Dame-de-Lorette, situés dans le Pas-de-Calais, sont des sites de mémoire. Le président Macron, comme chaque Président de la République au cours de son mandat, s'est rendu à Ablain-Saint-Nazaire sur la tombe des 45 000 soldats morts lors de la Première Guerre mondiale. Sur l'Anneau de la mémoire sont rassemblés rien de moins que 600 000 noms de soldats tombés dans le Nord-Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Je suis originaire de ce village et j'ai compris très vite, enfant, combien la paix est fragile, que rien n'est jamais acquis, qu'il ne faut rien oublier. Les manifestations patriotiques sont une occasion de comprendre qu'un pays a une histoire et un passé rempli de sacrifices- le présent, Il faut combattre la guerre, mes chers amis. La mort de milliers d'êtres humains est toujours une tragédie, quelle que soit l'époque. Rechercher l'entente entre les nations doit être la priorité avant de tomber dans l'irréparable. L'année 2018 a été une année historique d'anniversaire et de transmission. Si nous comprenons parfaitement qu'une partie des crédits affectés à la commémoration du centenaire de la Grande Guerre n'aient pas été reconduits au titre des années suivantes, nous avions déjà constaté, l'année dernière, une baisse de 2,79 millions d'euros des crédits qui n'avait rien à voir avec la fin de la

Un sondage récent indiquait que 25 % des Français de 18 à 25 ans ne savaient pas ce qu'était l'Holocauste ! Nous ne pourrons faire face à de tels fléaux que par la transmission des valeurs républicaines et patriotiques. La politique de mémoire est donc indispensable, et je regrette sincèrement cette baisse des crédits. Investir dans le devoir de mémoire est une évidente nécessité pour former les citoyens de demain. La baisse continue des crédits affectés à cette politique démontre que la transmission des valeurs patriotiques n'est pas une priorité du moment. J'ai malgré tout envie de croire dans le succès futur du service national universel obligatoire,

et après réflexion, je préfère voir le verre à moitié plein. Je voterai donc les crédits de la mission. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, honorer nos combattants, honorer leur engagement, honorer leur mémoire, nous le faisons lors des différentes manifestations patriotiques

Madame la secrétaire d'État, les budgets relatifs aux anciens combattants se suivent et se ressemblent : ils sont en baisse régulière. La diminution pour 2020, de l'ordre de 6,2 %, est une nouvelle fois justifiée par la baisse naturelle du nombre des bénéficiaires, mais surtout par la rigueur budgétaire.

Dans ce contexte budgétaire, l'année 2019 a vu la mise en place d'une mesure maintes fois réclamée, elle aussi, dans cette assemblée, à savoir l'extension de la carte du combattant : 35 000 cartes devraient être attribuées en 2019. Cette réussite a été rendue possible grâce à la mobilisation des associations d'anciens combattants, de l'ONAC-VG et de son réseau de proximité. C'est l'occasion, aujourd'hui, de les remercier. depuis votre prise de fonction et dans le cadre de la feuille de route que vous nous aviez présentée en 2018, vous avez engagé un temps de concertation avec les grandes associations sur toutes les questions qu'elles souhaitent voir traiter ; mais elles attendent désormais des avancées significatives, car seule, à ce jour, depuis votre prise de fonction, l'extension de la carte du combattant a été prise en compte. Concernant le budget pour 2020, vous avez tenu à maintenir l'ensemble des dispositifs de reconnaissance et de réparation au profit des anciens combattants. Vous avez tenu à prévoir plusieurs mesures au profit des personnes vulnérables : une augmentation de la pension militaire d'invalidité des conjoints survivants de grands invalides de guerre ayant passé auprès d'eux plus de dix ans de soins constants le maintien des crédits d'action sociale au niveau qui est le leur depuis plusieurs années, en dépit de la diminution du nombre de ressortissants ; la revalorisation de l'allocation de reconnaissance bénéficiant aux anciens harkis et la mise en place d'un fonds de solidarité au profit de leurs enfants en difficulté. On peut toutefois regretter

et victimes de guerre (UDAC) des Deux-Sèvres ont réuni les parlementaires du département pour faire le point sur le projet de budget pour 2020. Ils demandent depuis longtemps que la valeur du point servant de base de calcul pour plusieurs dispositifs puisse être actualisée et redéfinie. et redéfinie. Vous aviez d'ailleurs donné votre accord pour l'installation d'une commission tripartite chargée d'évaluer l'impact du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations. Pouvez-vous nous confirmer qu'une telle commission sera bien mise en place en 2020 ? Ils demandent également que le bénéfice de la campagne double soit attribué en fonction du temps passé sur un territoire de guerre, et non plus en fonction des actes de feu. Ils demandent que soit accordé le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire aux veuves dont le mari est décédé avant 74 ans. Ils demandent la revalorisation de la retraite du combattant- la dernière augmentation date du 1 septembre 2017. Ils demandent enfin le maintien des offices départementaux en tant qu'échelon de proximité. Ils craignent en effet que la réorganisation des services de l'État ne fasse évoluer également l'organisation des offices sur notre territoire.

En conclusion, madame la secrétaire d'État, vous le savez, le monde des anciens combattants ne demande pas de récompense ; il demande seulement un droit à la reconnaissance et une réparation qui s'impose. Nous comptons sur vous pour ne pas le décevoir ! La parole

ce jour de présentation devant vous du budget relatif au monde combattant et au lien entre l'armée et la Nation est un jour particulier- vous l'avez tous noté. Il suit une journée très difficile pour notre ministère des armées, mais aussi pour la France, avec la disparition tragique, au Mali, au cours de combats contre des terroristes, de treize soldats français. Je veux à mon tour, devant vous, rendre hommage à ces combattants, à ces héros morts pour la France, à leur engagement sans faille pour protéger notre pays. Je veux avoir une pensée émue pour toutes leurs familles, qui sont si éprouvées, et une pensée particulière, ici, au Sénat, pour Jean-Marie Bockel, votre collègue et ami, mais aussi un de mes prédécesseurs en charge du monde combattant ; je veux lui dire toute mon affection et tout mon soutien. Je veux dire aussi notre solidarité avec tous nos soldats, toutes ces femmes et tous ces hommes qui assurent notre sécurité et notre liberté. Le monument aux morts pour la France en opérations extérieures inauguré le 11 novembre dernier par le Président de la République permettra de rappeler à tous les Français l'intensité permanente de cet engagement, et aux familles de savoir la reconnaissance de la Nation et de se recueillir ; il nous permettra à tous d'honorer nos héros. Les symboles et les monuments de notre mémoire nationale sont malmenés depuis quelques mois ; ils l'ont été récemment encore, place d'Italie, ici, à Paris. Outre mon indignation, je veux redire que le lien entre l'armée et la Nation est un guide essentiel pour notre communauté nationale et pour sa cohésion que ce lien est indissociable de la reconnaissance et du respect de tous envers nos anciens combattants et nos combattants d'aujourd'hui ; qu'il doit être entretenu par un travail de mémoire actif et qu'il doit être développé auprès de la jeunesse de France. C'est l'ambition que je porte avec le projet de budget que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Ce budget pour 2020 est à la fois un budget de continuité, de pérennisation et d'évolution. Continuité, car tous les droits des anciens combattants sont préservés. Tous ! Pérennisation, avec la traduction budgétaire de la montée en puissance de l'attribution de la carte du combattant « 62-64 »

Pérennisation et évolution, afin de toujours mieux prendre soin des personnes les plus vulnérables- j'ai fait de ce sujet un axe majeur des politiques que je souhaite mener auprès du monde combattant. Nous maintenons à 26 millions d'euros la dotation d'action sociale de l'ONAC-VG malgré la diminution du nombre de ses ressortissants. Nous majorons les pensions militaires d'invalidité versées aux conjoints survivants d'un grand invalide de guerre présents à leur côté pendant de nombreuses années- ces aidants sont remarquables. Pérennisation des missions de l'Office national des anciens combattants, opérateur essentiel pour le monde combattant, et pérennisation de son ancrage départemental. Oui, l'ONAC-VG va évoluer par ses modes opératoires et va s'adapter à l'évolution du monde combattant pour mieux servir.

2,5 millions d'euros d'économies se traduiront par une organisation territoriale qui s'adaptera à l'évolution du monde combattant. Ces mesures ont été votées à l'unanimité par le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants. Vous pouvez être assurés de notre volonté

Pérennisation de notre engagement fort auprès de l'Institution nationale des invalides (INI), en fonctionnement, bien sûr, mais aussi en investissement : 13,5 millions d'euros seront consacrés en 2020 à de lourds travaux d'infrastructure qui démarreront en janvier prochain. Nous voulons accompagner cet établissement dans son évolution vers un grand pôle de réhabilitation physique et psychique pour nos blessés. À cet égard, je viens de signer une convention de partenariat entre le service de santé des armées et l'INI, convention qui vise à créer ce grand pôle de réhabilitation post-traumatique de défense. C'est une avancée concrète pour la prise en charge des blessés et des anciens combattants. Le budget « mémoire » est consolidé 11 millions d'euros de dotations budgétaires, auxquelles s'ajoute un prélèvement à hauteur de 4 millions sur la trésorerie de l'ONAC, toujours de manière exceptionnelle. L'effort sera fait sur l'entretien et la réhabilitation des hauts lieux de mémoire et des sépultures, sur la préparation des thématiques mémorielles de 2020, qui sera l'année du général de Gaulle,

de les consacrer à la lutte contre la haine et les préjugés en cette année 2020 où nous célébrerons le soixante-quinzième anniversaire de la libération des camps de concentration. Enfin, un effort est fait sur les crédits consacrés au lien entre les armées et la jeunesse. Le service militaire volontaire est pérennisé dans son fonctionnement dans la loi de programmation militaire.

La Journée défense et citoyenneté sera bien sûr progressivement remplacée par la montée en puissance du service national universel. En conclusion, c'est un budget global de 2,16 milliards

Ce budget respecte tous les engagements pris au fil des législatures en termes de reconnaissance et de réparation. C'est un budget qui prend soin des plus fragiles et qui continue à tisser le lien indispensable entre l'armée et la Nation. C'est un budget réaliste, sincère, volontariste. Il met en oeuvre des mesures qui étaient très attendues depuis de nombreuses années. Je pense à la mesure « 62-64 » : c'est un engagement qui a été honoré. Je continuerai, bien sûr, à travailler avec les associations, en suivant la méthode que je leur avais proposée lorsque j'ai pris mes fonctions. sur des groupes de travail qui nous permettent d'avancer ensemble toujours plus, pour reconnaître ce monde combattant, pour l'accompagner et surtout pour lui dire au quotidien le respect que nous lui portons, ainsi qu'aux familles, aux veuves et aux enfants.

Deux points, car il s'agit de renouer avec la dynamique en faveur des anciens combattants instaurée entre 2005 et 2012. La majorité des bénéficiaires sont âgés, certains d'entre eux sont fragiles, d'autres sont dans la précarité et d'autres encore sont dans des situations de dépendance. Ils méritent des conditions de vie décentes. La Nation doit manifester cette reconnaissance concrètement, justement et décemment. Le coût s'établit à 18 millions d'euros en année pleine et le financement peut se faire par l'action n° 01, Liens armées-jeunesse, On pourrait me faire le reproche de prendre sur des moyens consacrés aux jeunes. Mais en réalité, je souhaite vivement que les budgets et dispositifs existants- la JDC et le SMV -fassent l'objet d'une évaluation et d'une répartition entre les ministères concernés. Au moment où le Gouvernement expérimente un service national universel, financé à hauteur de 30 millions d'euros sur la mission « Sport, jeunesse et vie associative », il est temps de s'interroger sur la pérennité des financements de la JDC au regard des objectifs depuis sa création. Force est de constater que les contextes sécuritaire et civique ont profondément évolué. La mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » finance la JDC à hauteur de 15,6 millions sur un total de 106,2 millions. Le SNU représente donc le double des crédits de la JDC au sein de cette mission. Ce qui doit nous préoccuper, c'est l'efficacité des différents dispositifs. Nous considérons aujourd'hui que la priorité budgétaire est de revaloriser la retraite des combattants.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à pallier une inégalité dans notre dispositif d'indemnisation des orphelins de parents victimes d'actes de barbarie ou d'actes de persécution, tel qu'il est défini par le décret du 13 juillet 2000, qui exclut de fait les pupilles de la Nation. Ces enfants dont les parents résistants sont morts pour la France les armes à la main, avec la mention « mort pour la France » sur les registres d'état civil, restent des orphelins de la Seconde Guerre mondiale. Plus de soixante-dix ans après la fin de ce conflit, il est temps, dans un travail de mémoire, de ne plus faire de différence entre les victimes de la Seconde Guerre mondiale.

pas favorable. Je rappelle que la retraite du combattant a été réévaluée chaque année entre 2006 et 2012 de 1 point, puis de 4 points en 2017. Elle a été portée de 33 à 52 points.

Cette année, j'ai fait le choix d'apporter un soutien supplémentaire aux plus fragiles, mais j'ai également décidé de répondre au souci décidé de répondre au souci des associations en mettant en place une commission tripartite, que vous avez les uns et les autres évoquée dans vos propos introductifs. Cette commission tripartite réalisera une étude sur l'évolution du point de PMI par rapport à l'inflation.

Elle permet de renforcer la cohésion nationale et l'insertion sociale des jeunes en difficulté. Ce dispositif est de niveau législatif et il nous est impossible de diminuer ce budget.

Gouvernement ? Le décret de 2000 a créé un dispositif d'indemnisation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Puis, le décret de 2004 a créé un dispositif identique pour les orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie, déportés résistants ou politiques. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle, qui est de consacrer solennellement

: La parole est à Mme Sabine Van Heghe. Nous souhaitons soutenir et encourager le dispositif du service militaire volontaire, créé à titre expérimental en 2015, puis définitivement mis en place par la loi du 13 juillet 2018. Ce dispositif, inspiré de celui que l'on trouve dans les outre-mer, a montré son efficacité et s'est bien implanté dans l'Hexagone. Pour les premières promotions, le taux d'insertion professionnel a même dépassé les 74 %, ce dont nous nous réjouissons. Toutefois, Toutefois, alors que le Gouvernement indique que le SMV a reçu 1 200 jeunes en 2019 et que 300 de plus devraient venir en étoffer les rangs en 2020, le « bleu » budgétaire mentionne quant à lui un budget réduit. Effectivement, là où 1 500 jeunes seront reçus, les crédits alloués ne suffisent que pour 1 000 Se pose alors la question de l'insuffisance des moyens mis en place à laquelle nous souhaitons apporter une réponse financière, afin d'offrir à ces jeunes la possibilité d'évoluer dans des conditions optimales. Le budget pour 2020 étant identique à celui de 2019, nous proposons logiquement, par le biais de cet amendement, d'augmenter les moyens dévolus au SMV

La baisse du nombre de ressortissants n'est pas une raison pour comprimer le budget de l'ONAC-VG comme vous le faites. Entre 2012 et 2017, nous avions augmenté chaque année de 1 million d'euros le budget de l'action sociale de l'ONAC-VG, et ce malgré la baisse du nombre de ressortissants, pour le porter de 21 millions à 26 millions d'euros. Depuis, ce budget ne retrouve malheureusement pas son souffle. Pourquoi devons-nous augmenter les crédits de l'ONAC-VG ? D'une part, l'ONAC-VG doit faire face aux surcoûts liés à la gestion opérationnelle du plan en faveur des rapatriés et des harkis. D'autre part, l'élargissement de la carte du combattant aux soldats engagés entre 1962 et 1964 a donné lieu à la délivrance de 35 000 cartes supplémentaires. Par ailleurs, l'accompagnement des veuves non imposables d'anciens combattants constitue également une charge de travail importante, qui relève de cet organisme. Enfin, la prise en charge psychologique et financière des victimes du terrorisme, qui est l'une des nouvelles missions de cet office, ne s'essoufflera malheureusement pas. C'est notamment pour faire face à tous ces éléments que nous souhaitons voir le budget de l'ONAC-VG augmenter. Quel

Vous avez également parlé d'actions sociales. L'action sociale est maintenue à 26 millions d'euros et la subvention pour charges de service public

nous avons le regret de constater aujourd'hui que le soutien aux projets mémoriels perd 540 000 euros. Le budget consacré aux actions pédagogiques reste inchangé, à hauteur de 350 000 euros, alors même que les associations d'anciens combattants n'ont eu de cesse de rappeler l'importance de développer ces actions auprès de nos jeunes.

nous avons consacré 350 000 euros aux actions pédagogiques réalisées par le ministère et prévu 150 000 euros qui sont délégués à l'ONAC-VG.

Actions en faveur des rapatriés, du programme 169, « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ». La Nation a un devoir de justice envers les membres de nos forces supplétives en Algérie, quel que soit leur statut. Le présent amendement vise à régler définitivement la situation des membres rapatriés de nos forces supplétives de statut civil

local. Cette différenciation a été validée juridiquement par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ont mis en avant le droit à l'allocation de reconnaissance, qui a été ouvert de façon temporaire et

ces personnes ont fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'administration, non suivie de recours contentieux. Dans leur cas, le refus de l'administration est donc devenu définitif.

d'essayer de régler humainement cette situation. J'ai ainsi chargé l'ONAC-VG de contacter ces personnes afin de savoir si elles souhaitaient bénéficier d'une aide sociale. Sur les 24 personnes contactées, 3 sont décédées, 15 n'ont pas souhaité donner suite à cette proposition et 6 ont effectué une demande de secours ; parmi ces dernières, 2 ont déjà reçu une aide importante. Enfin, un dossier est encore en cours d'étude.

puis de nouveau de 0,6 % en février 2017 -, les précédentes revalorisations du point de PMI n'ont pas réussi à effacer les pertes de pouvoir d'achat. La valeur du point de PMI servant au calcul du montant des pensions militaires d'invalidité

retard du point de PMI et de définir les moyens de le combler, avec l'objectif de préparer une prochaine revalorisation devant s'opérer par la voie réglementaire. Quel

Il permet de revaloriser les pensions militaires plusieurs fois par an, chaque fois que l'indice évolue, et de façon rétroactive. La valeur de ce point continuera à augmenter de 2019 à 2021, du fait de la poursuite de l'entrée en vigueur du protocole relatif aux parcours professionnels,